La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 3 octobre 2018 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? Le procès-verbal est adopté. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

ait retenu ce régime de responsabilité solidaire des plateformes. Je le répète, un projet de loi relatif à la lutte contre la fraude qui aurait omis la fraude à la TVA sur internet aurait été très incomplet. Ne l'oublions pas, l'article 4 du projet de loi, relatif à l'obligation de déclaration automatique des revenus par les plateformes,

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs,

J'y vois la preuve que son ambition, à savoir la modernisation de nos outils de lutte contre la fraude pour les adapter aux fraudes du XXI siècle, fait l'objet d'un large consensus de la part de la représentation nationale. Aussi cette tribune sera-t-elle pour moi l'occasion de redire l'ampleur du travail mené par le Sénat, en particulier par son rapporteur, pour y parvenir. De fait, la discussion parlementaire a considérablement enrichi le texte présenté par le Gouvernement, qui comportait onze articles. Le Sénat en a ajouté dix-huit, dont l'Assemblée nationale a conservé la moitié, concernant notamment la répression du délit de blanchiment douanier, les obligations déclaratives pour les comptes détenus à l'étranger, l'extension de la convention judiciaire d'intérêt public à la fraude fiscale, la lutte contre les trafics sur le tabac ou encore le rétablissement de la faculté transactionnelle de l'administration fiscale en cas de poursuites pénales. Ces apports majeurs ont largement contribué à ce qu'un accord soit trouvé entre les deux chambres.

que l'Assemblée nationale a souhaité renforcer par un alignement des prérogatives des officiers fiscaux judiciaires sur celles des officiers des douanes judiciaires. De la même manière, je me réjouis du pragmatisme dont a su faire preuve le Sénat s'agissant de la réforme de la procédure pénale applicable à la fraude fiscale, autrement dit du « verrou de Bercy De ce point de vue, l'Assemblée nationale a utilement complété le travail de votre rapporteur en définissant précisément les critères objectifs de gravité conduisant à une dénonciation automatique des dossiers au parquet. Surtout, l'article 13 tel qu'il est issu de vos travaux permettra indéniablement une meilleure collaboration entre l'autorité judiciaire et l'administration fiscale, comme cela se pratique dans nombre de pays. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet, si vous le souhaitez, pour vous présenter la circulaire d'application que la garde des sceaux, Gérald Darmanin et moi-même sommes en train de préparer. Je me Je me réjouis par ailleurs que le Sénat accueille avec bienveillance plusieurs apports bienvenus nés du dialogue entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale. Je pense ici aux initiatives conjointes des groupes communistes, socialistes, Modem et France insoumise, afin de prévoir à l'article 11 la possibilité d'inclure des États de l'Union européenne dans la liste des États et territoires non coopératifs. J'évoquerai également un autre article, issu d'un amendement déposé par le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, pour moderniser la procédure d'autorisation d'accès aux données de connexion par l'Autorité des marchés financiers, la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects. mixte paritaire est également pour moi l'occasion de saluer les avancées obtenues dans ce texte concernant les plateformes d'économie collaborative. Je sais l'attachement de votre assemblée, en particulier de votre commission des finances, à une meilleure appréhension de la fraude susceptible d'en résulter. Je pense tout d'abord à l'article 4, qui précise, comme le Parlement y invitait le Gouvernement depuis plusieurs années, les obligations fiscales et sociales imposées aux plateformes d'économie collaborative. J'évoquerai également l'article 4 , qui prévoit, à compter de 2020, un régime transitoire de responsabilité solidaire des plateformes en matière de TVA due par les vendeurs et prestataires, dans l'attente de la transposition de la directive adoptée à Bruxelles en fin d'année dernière. Concrètement, lorsqu'existent des présomptions qu'une personne se livrant à des activités en France par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de TVA, TVA, l'administration pourra mettre en demeure l'opérateur de la plateforme de prendre les mesures permettant à la personne en cause de régulariser sa situation. En l'absence de régularisation, la plateforme est solidairement tenue au paiement de la TVA due par cette personne. Il s'agit d'une avancée majeure, qu'il Enfin, le texte issu de la commission mixte paritaire démontre utilement, me semble-t-il, la vigilance dont a su faire preuve le Sénat, pour conjuguer lutte contre la fraude et pragmatisme économique. Cela permet que notre détermination absolue à lutter contre ce phénomène ne se fasse pas au détriment de la compétitivité de notre économie. Vous me permettrez ici de donner trois exemples.

aux personnes morales et en ajoutant l'obligation de publier toute décision contentieuse favorable au contribuable, lorsque celle-ci intervient après la publication des résultats d'un contrôle ayant donné lieu à redressement et sanctions.

à une condamnation pénale ou à une sanction définitive du contribuable abusivement conseillé. Je me réjouis, à la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire, que cette disposition, qui aurait privé la mesure de toute efficacité et l'aurait détournée de son objectif, n'ait pas été retenue. Rappelons-le, cet article n'a pas pour objet dissimulé de mettre à mal la profession d'avocat ni celle d'expert-comptable. Il ne constitue pas une atteinte au secret professionnel, ce dernier restant applicable, sauf si le client le lève. En réalité, cet article vise non pas tant les professions réglementées, qui disposent déjà de leurs propres règles déontologiques, que toutes les officines qui, en dehors de tout cadre réglementé, fournissent des solutions pour échapper purement et simplement à l'impôt. La liste des prestations donnant lieu à sanction, définies dans cet article de façon restrictive, rassure tous ceux qui exercent leur profession de conseil honnêtement : ils pourront continuer à le faire sans crainte d'être inquiétés. Dernier exemple : la commission mixte paritaire a fait preuve de pragmatisme en choisissant de conserver l'amendement de l'Assemblée nationale qui prévoit d'élargir le contenu du rapport extrafinancier des entreprises cotées, pour qu'il aborde également la lutte contre l'évasion fiscale, mais en supprimant l'obligation de communiquer aux représentants du personnel la documentation sur les prix de transfert, qui restera bien évidemment à la disposition de l'administration en cas de contrôle fiscal. Mesdames, messieurs les sénateurs, la lutte contre la fraude est un objectif que nous partageons tous- cela a été rappelé tout au long des débats. Son ampleur est immense, mais nous avons la faiblesse de croire que, en dotant l'administration et la justice de nouveaux outils adaptés aux fraudes actuelles, ce texte contribuera à lutter contre des comportements frauduleux de plus en plus retors et dangereux. La contribution de votre assemblée à son enrichissement a été décisive. Je me réjouis de son adoption par la commission mixte paritaire.

en ces jours de commémoration du soixantième anniversaire de la Constitution de la V République, j'ai envie de faire référence à Georges Pompidou. Très bien ! Ce dernier évoquait déjà durant les trente glorieuses le fléau de la fraude fiscale : « La fraude est à l'impôt ce que l'ombre est à l'homme. Les propos de l'ancien Président de la République n'ont jamais cessé d'être d'actualité. Nous y répondons aujourd'hui par un texte que l'on pourrait qualifier de « bélier », fruit d'un débat parlementaire riche, qui illustre bien, s'il le fallait encore, que le bicamérisme est un impératif démocratique pour notre pays. Je me réjouis que la commission mixte paritaire, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer en tant que représentante du groupe du RDSE, soit parvenue à l'adoption d'un texte commun. Après la promulgation cet été de la loi pour un État au service d'une société de confiance, ce texte représente le volet « répressif » des nouvelles relations entre l'État et les citoyens que le Gouvernement souhaite engager. Son objet est simple : permettre de mieux détecter, de mieux appréhender et de mieux sanctionner les différentes formes de fraude, qui sont autant d'entorses à notre contrat social. le rappelle, la fraude fiscale coûte entre 60 milliards et 80 milliards d'euros par an, soit près de 20 % des recettes fiscales brutes de notre pays. Ce sont autant de ressources en moins pour financer les politiques publiques et réduire nos déficits. Ce sont autant d'efforts en plus que nous demandons à nos concitoyens pour combler ce manque à gagner. L'examen parlementaire a considérablement enrichi le texte du Gouvernement, qui, de onze articles dans sa version initiale, est passé à En tant que rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, j'avais proposé en première lecture, conformément à l'avis du Conseil d'État, la suppression de l'article 1, auquel faisait référence M. le rapporteur. apparaissait en effet redondant avec les dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale au sein du ministère de l'intérieur. Je comprends la nécessité pour la commission mixte paritaire de parvenir à un compromis, mais je regrette le maintien de cet article, qui revient à créer un nouveau service de police fiscale au sein du ministère des comptes publics, à côté de la brigade nationale de répression de la délinquance financière. Cela risque de se traduire, au mieux, par un jeu à somme nulle, au pire, par une guerre des polices. Je salue en revanche le maintien de l'article 9 que j'avais défendu. Il concerne la convention judiciaire d'intérêt public, une « transaction pénale » ouverte en matière de fraude fiscale. Ce nouvel outil permettra de renforcer l'efficacité des modes de poursuite, tout en assurant la publicité et la transparence pour ce qui concerne la fraude effectuée. Je regrette toutefois que les députés aient supprimé l'article 9 qui aurait permis d'inscrire dans la loi la jurisprudence, laquelle précise que le « verrou de Bercy » ne s'applique pas au délit de blanchiment de fraude fiscale.

je conçois parfaitement que notre droit évolue en ce sens pour les seules personnes morales, étant entendu que la fraude fiscale a atteint un degré d'acceptabilité sociale particulièrement bas. C'est également le sens qu'il faut donner à l'évolution des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers en matière de lutte contre les abus de marché, adoptée par la commission mixte paritaire. Il s'agit d'anticiper une inconstitutionnalité qui devait prendre effet à la fin de l'année. J'en viens à la réforme du « verrou de Bercy », point majeur de ce texte, auquel les médias ont consacré une attention peut-être disproportionnée au regard des autres dispositions. Il est revenu à la Haute Assemblée de poser les bases du débat, de façon transpartisane, en instaurant des critères rendant obligatoire la transmission au parquet des dossiers de fraudes fiscales les plus graves, supérieures à 100 000 euros. L'Assemblée nationale a complété notre texte en renforçant le dispositif et la gravité des sanctions, notamment pour les élus.

À l'échelle internationale, l'accord multilatéral de 2016 sur l'échange de déclarations pays par pays et la convention multilatérale de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, ratifiée par la Haute Assemblée le 19 avril dernier, ont représenté une petite avancée. aujourd'hui n'est pas encore exemplaire dans son aboutissement, il est significatif. C'est à ce titre que mon groupe le soutiendra et votera en faveur de l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire. La parole

je tiens en préambule à féliciter les rapporteurs, qui ont contribué à l'aboutissement de ce texte. Ses avancées sont nombreuses et significatives. Les discours sur la répression de la fraude fiscale ont souvent été incantatoires, faute d'être accompagnés, comme il se devait, par un renforcement de l'arsenal législatif. Animés ici d'un même volontarisme politique visant à réprimer les comportements frauduleux et, ce faisant, consolider le pacte fiscal et social qui relie entre eux chacun de nos concitoyens, Sénat et Assemblée nationale sont intelligemment parvenus à trouver des compromis sur les quarante-trois articles qui restaient encore en discussion. Ça arrive ! Le groupe Union Centriste se réjouit de l'issue conclusive de cette commission mixte paritaire. Le Sénat aura pesé de tout son poids dans la discussion, démontrant une nouvelle fois par la rigueur de ses travaux et la qualité de son expertise à quel point il est indispensable à la vitalité du débat démocratique. Certes, nous pouvons déplorer la suppression par l'Assemblée nationale de neuf des dix-huit articles additionnels insérés par la Haute Assemblée. Mais nous pouvons surtout nous satisfaire de l'adoption en termes identiques de nombreuses dispositions,

en cas de poursuites pénales, ou encore du rétablissement de l'article 6 dans la rédaction adoptée par le Sénat, qui permet d'écarter les personnes physiques du dispositif de publication des sanctions, en parfaite conformité avec le droit au respect de la vie privée. Le Sénat aura globalement veillé à garantir la sécurité juridique et l'efficacité des régimes de sanctions et des procédures fiscales contenues dans le projet de loi. comment ne pas se féliciter du rétablissement de l'article 4 qui introduit un régime de responsabilité solidaire des plateformes en ligne en cas de non-paiement de la TVA par les vendeurs ? La commission des finances du Sénat et son rapporteur général l'ont souligné : depuis que nos voisins Britanniques ont mis en place ce système, la fraude à la TVA sur internet a reculé, tandis que les recettes fiscales afférentes à cet impôt ont augmenté. L'enjeu n'est pas mince, mes chers collègues, la TVA fournissant à elle seule la moitié des recettes budgétaires de l'État. J'aimerais enfin saluer l'action décisive du Sénat s'agissant du « verrou de Bercy

Réserver un traitement différencié pour les élus et hauts fonctionnaires, comme certains l'exigeaient, eût été fouler aux pieds les principes constitutionnels les plus élémentaires. Si nul ne doit être au-dessus de la loi, la réciproque est aussi vraie : nul ne doit être en dessous L'État de droit nous fournit un cadre solide et exigeant où affichage et démagogie politiques n'ont pas leur place. Grâce à l'implication constructive de chacun,

nous sommes heureux que la CMP ait abouti à un accord. C'est suffisamment rare, par les temps qui courent, pour être souligné. Eh oui ! C'est le signe que nos deux assemblées peuvent se retrouver sur des positions communes, au service de l'intérêt supérieur de la Nation. fait, y a-t-il un intérêt supérieur à celui de s'assurer que l'impôt, qui se trouve au coeur du lien civique, est levé conformément à la loi ? Nous touchons ici au coeur de l'État. Le texte issu de la CMP est sensiblement différent du texte d'origine. Il est d'abord beaucoup plus important, puisqu'il a triplé de volume. Nous qui nous interrogeons sur la façon de mieux légiférer, convenons qu'il y a là, peut-être, un peu d'inflation législative Il a également été le support d'une réforme d'envergure. Cela a été évoqué, le « verrou de Bercy » est considérablement desserré, sur l'initiative du législateur. Beaucoup de fantasmes entourent cette procédure, qui n'avait pourtant qu'un but : rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire faciliter le recouvrement des sommes dues par le fraudeur à l'administration fiscale. La tentation était grande- et certains y ont succombé -de voir dans l'autorité judiciaire un parangon de vertu et dans l'administration le bras armé du copinage et du renoncement.

Ne pas fixer de seuil pour le montant des droits éludés pour les seuls élus et fonctionnaires aurait ainsi posé une sérieuse question de constitutionnalité. Je félicite M. le rapporteur d'avoir proposé de fixer un seuil égal à la moitié du montant prévu pour les autres contribuables. Cela me paraît plus raisonnable et parfaitement compréhensible par nos concitoyens. Pour ce qui concerne les autres sujets abordés par ce projet de loi, plusieurs dispositions me semblent aller dans le bon sens. Le voulu par le Gouvernement, s'il est utilisé avec mesure et à propos, peut être un outil redoutable dans la lutte contre la fraude. La commission mixte paritaire a fait preuve de discernement devant le texte proposé par l'Assemblée nationale. Un amendement du groupe La France insoumise étendait cette publicité aux personnes physiques cette disposition était manifestement incompatible avec le droit au respect de la vie privée, protégé par des principes constitutionnels et issu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La proposition de la CMP de publier des décisions qui donnent raison au contribuable est la bienvenue, car elle renforce les garanties de la procédure. Je me félicite également que le Sénat ait obtenu gain de cause au sujet de la fraude à la TVA sur les plateformes en ligne. L'instauration d'une responsabilité solidaire des plateformes est une proposition récurrente de notre commission des finances. Elle complètera utilement la prochaine directive TVA, qui entrera en vigueur en 2021. Enfin, la suppression de l'inscription de la jurisprudence dans le texte évitera d'ouvrir une boîte de Pandore au préjudice de la sécurité juridique. Les magistrats y étaient eux-mêmes opposés, tant sa légalisation présentait plus d'inconvénients que d'avantages. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants - République et territoires se félicite qu'une position de compromis ait pu être trouvée sur ce texte, qui se prêtait à tous les excès et à toutes les caricatures. La lutte contre la fraude fiscale est un objectif de première importance, mais elle ne doit pas conduire à éluder d'autres principes tout aussi importants : respect de la présomption d'innocence et des libertés individuelles, nécessité de recouvrer l'impôt, équilibre entre le rôle de l'administration et celui du juge ... La tentation est grande, en matière de morale, de vouloir déchaîner l'appareil administratif et judiciaire contre les fraudeurs.

que c'est la force de notre République de punir avec justice et mesure, de prévenir avec fermeté et efficacité, de légiférer avec tempérance et souci de l'intérêt collectif. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je ne peux que le souligner et l'approuver.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, l'Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus à un accord sur un texte important pour

Ce texte est important parce qu'il intervient comme une réponse pragmatique à une question clé dans le respect de notre pacte républicain. Gardienne d'un temps long au bénéfice de l'intérêt général, notre assemblée doit se réjouir de mesures qui n'ont été prises ni dans l'émotion ni dans la réaction. La fraude fiscale bafoue nos principes républicains les plus essentiels. Elle mine les finances publiques, à hauteur de 30 milliards à 80 milliards d'euros selon les années- autant d'argent non investi au service des Françaises et des Français.

Elle a conservé des ajouts utiles du Sénat, comme la répression du délit de blanchiment douanier, les obligations déclaratives pour les comptes détenus à l'étranger, l'extension de la convention judiciaire d'intérêt public en matière de fraude fiscale, la lutte contre les trafics sur le tabac ou encore le rétablissement de la faculté transactionnelle de l'administration fiscale en cas de poursuites pénales. Je veux revenir sur les points principaux du texte final.

D'une part, les agents de la police fiscale disposeront, pour l'accomplissement de leurs missions, des mêmes pouvoirs que les officiers de police judiciaire ou des douanes judiciaires. D'autre part, cette police fiscale est un moyen supplémentaire de lutte contre la fraude : ni les moyens de la brigade nationale de répression de la délinquance me semble-t-il, l'objectif essentiel de ce projet de loi : apporter des réponses pragmatiques à des comportements frauduleux. L'article 2 renforce les moyens de lutte des agents des douanes contre les logiciels conçus pour permettre ou organiser la fraude. Cette mesure de bon sens répond à un besoin des agents des douanes. Le projet de loi rend par ailleurs plus effectif le droit de communication, au bénéfice de la recherche de la fraude douanière et de l'établissement de l'assiette des impositions douanières. Tout aussi

équilibré en ce qu'il dispense de l'obligation de transmission les plateformes dont les revenus sont exonérés par nature, comme celles de mise en relation pour du covoiturage ou de publication d'annonces pour la vente de biens d'occasion entre particuliers,

Ce texte est pragmatique, mais il n'est pas que cela. En réalité, le pragmatisme et l'exemplarité en sont les deux caractères. Je pense à l'introduction du en droit français, à l'article 6, ou encore à l'automaticité de la peine complémentaire de publication en cas de fraude fiscale. Ce sont là deux mesures

l'article 13, relatif au verrou de Bercy, tant il tient une place importante dans le texte issu des travaux du Sénat et de l'Assemblée nationale. Durant les dernières décennies, le sujet du verrou de Bercy a été régulièrement évoqué, quelle que soit la majorité

dispositif proposé par notre collègue députée Émilie Cariou est simple : l'administration devra informer le parquet des manquements fiscaux au-delà de 100 000 euros de droits rappelés et ayant donné lieu aux pénalités les plus importantes- 100 % et 80 % ou 40 % en cas de réitération. Ces critères sont assortis d'une souplesse pour l'administration fiscale, qui pourra transmettre les dossiers n'y répondant pas strictement. Par ailleurs, l'avis préalable de la commission des infractions fiscales pour les dossiers de présomption caractérisée est supprimé. L'administration pourra ainsi déposer plainte directement pour ces dossiers de suspicion de fraude fiscale, ce qui permettra au parquet d'étendre plus rapidement ses investigations lorsqu'il découvrira une fraude fiscale connexe à une infraction sur laquelle il enquête déjà. Mes chers collègues, je salue une nouvelle fois

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au lendemain de l'ouverture du procès de la banque suisse UBS, ce projet de loi de lutte contre la fraude prend tout à coup un visage quelque peu pâlichon. En effet, ce procès de toutes les démesures illustre à nouveau l'ampleur et la complexité de l'industrie de l'évasion fiscale. À l'occasion des premières annonces relatives à ce texte, il fut fait grand cas de la création d'une police fiscale,

du présent projet de loi aurait dû être l'occasion de renforcer la protection des lanceurs d'alerte et de reconnaître leur rôle au sein des entreprises. La République devrait leur apporter son soutien et leur témoigner sa reconnaissance, leur action permettant à l'État de récupérer des sommes considérables. Le cas de l'UBS est aussi emblématique du fait qu'il s'agit d'une banque suisse. Ce projet de loi prévoyait une révision de la liste française des paradis fiscaux, qui comporte sept États : Brunei, Nauru, Niue, le Panama, les Îles Marshall, le Guatemala

a appris que le tribunal administratif fédéral de Saint-Gall, en Suisse, donnait raison à la banque UBS, qui refuse de répondre à la demande d'assistance administrative lancée par notre pays. A-t-on fait appel de cette décision, comme la loi nous y autorise ? Et l'on nous dit que la Suisse n'est plus un paradis fiscal la banque UBS a tenté d'obtenir une « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ». Sans succès. En 2016, la loi a institué un nouvel outil de négociation inspiré du système américain,

En 2017, HSBC, pour éviter un procès, toujours dommageable pour la réputation d'une honorable banque, a accepté de payer une amende de 300 millions d'euros, après avoir reconnu une fraude de 1,6 milliard d'euros À l'heure où nos concitoyens doutent de plus en plus de l'action publique et de son exemplarité, ne pensez-vous pas, mes chers collègues, que ces dispositifs sont de nature à accréditer l'idée que la justice n'est pas la même pour tous ? Selon que vous serez puissant ou misérable, disait le fabuliste Le déroulement de cette CMP nous laisse aussi un goût amer au regard de la suppression d'un amendement qui avait été adopté à l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement il est vrai. Cet amendement portait sur la délicate question des prix de transfert au sein des entreprises. Les représentants du personnel jouant un rôle essentiel dans le combat contre la fraude, l'évasion et l'optimisation fiscales,

Nous ne pouvons que déplorer que cet amendement ait été supprimé lors de la CMP, jeudi dernier. Il constituait, aux yeux de beaucoup, une réelle plus-value pour le texte et la marque d'une volonté forte d'avancer sur les questions de transparence. Cette suppression est un échec incompréhensible.

Ce débat eut lieu au Sénat au printemps dernier, sans réel succès, puis en juillet à l'Assemblée nationale. La lumière jaillit soudain : un nouvel amendement accepté par le Gouvernement allait être adopté et venir enfin supprimer, nous disait-on, le fameux verrou de Bercy.

Oui, le verrou est desserré, mais il n'est pas supprimé complètement. Avec l'adoption de cet amendement, le fisc sera obligé de transmettre les dossiers les plus graves à la justice, selon des critères inscrits dans la loi : montant fraudé supérieur à 100 000 euros,

Le nombre des dossiers fiscaux qui seront transmis de façon automatique à la justice pourrait doubler, passant d'un millier aujourd'hui à environ 2 000 demain. C'est oublier que 4 000 dossiers considérés par l'administration fiscale comme relevant de fraudes graves ... Ces avancées sont à prendre en compte, mais elles sont notoirement insuffisantes, timides, au dire de nombreux observateurs. Nous prenons acte de la création de sanctions contre les intermédiaires dans ce texte. De fait, on ne peut jamais s'évader sans un peu d'aide ... Cette proposition figurait d'ailleurs dans les rapports des commissions d'enquête. Nous prenons également acte de la clarification opérée concernant les plateformes de l'économie collaborative. nous restons très nettement sur notre faim. Le compte n'y est pas. Le déroulement de la CMP a été particulièrement éclairant et a permis de jauger la réalité des intentions. Aussi, au terme de ce débat parlementaire, nous ne pouvons nous associer aux conclusions de la commission, et nous émettrons un vote négatif

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, chers collègues, la lutte contre la fraude fiscale est un combat de longue haleine, qui nous mobilise régulièrement. C'est l'un des plus grands défis du moment que de trouver les moyens d'en finir avec ce fléau, qui nuit à l'équilibre du budget des États et contrevient au pacte social en vertu duquel chacun contribue à hauteur de ses moyens au financement des politiques publiques et de la solidarité nationale. nous nous félicitons qu'un texte traite de ce sujet, dans la continuité des lois de 2013 et de 2016, et nous notons avec satisfaction un certain nombre d'avancées,

Nous saluons également la mise à disposition de l'administration de Bercy de nouveaux outils tels que le, la responsabilité des intermédiaires ou la création de la police fiscale. Cependant, au-delà de ces avancées notables, indiscutables, ce projet de loi représente, à notre sens, une série d'occasions manquées.

Mais nous pensons que, malheureusement, l'objectif principal du Gouvernement en matière de politique fiscale est d'aider les entreprises coûte que coûte, quitte à réduire les dépenses sociales pour équilibrer le budget.

celles qui interviennent après de grands scandales et celles dont l'objet est de compenser une politique fiscale très avantageuse pour les plus favorisés. Manifestement, ce texte s'inscrit dans la seconde catégorie ; c'est pourquoi nous nous abstiendrons.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, madame la rapporteur pour avis, mes chers collègues,

Créée par la loi Sapin 2, cette convention permet de régler rapidement un litige par le biais d'une transaction entre le procureur de la République et la personne mise en cause, la transaction étant ensuite homologuée par un juge. Elle implique le versement au Trésor public d'une amende d'intérêt public et la mise en oeuvre d'un plan de mise en conformité sous la tutelle de l'Agence française anticorruption. Un tel dispositif Notre commission des finances peut se réjouir d'avoir su convaincre l'Assemblée nationale, ainsi que le Gouvernement, de lever enfin le verrou de Bercy. Le

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je ne vous parlerai pas de la vraie-fausse suppression du « verrou de Bercy ». En revanche, je voudrais attirer votre attention

donné la rédaction de l'article 8 du projet de loi, le juge pénal va maintenant être obligé de surseoir à statuer le temps que le juge de l'impôt, qui est souvent le juge administratif, fixe le montant des impôts fraudés ; désormais, en effet, l'amende pénale pour fraude fiscale sera proportionnelle au montant des impôts fraudés. Or la jurisprudence de la Cour de cassation impose que le juge pénal recherche et détermine avec exactitude le montant des impôts fraudés servant de base de calcul aux pénalités proportionnelles. Cela résulte notamment d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 1994, qui fait jurisprudence. En matière fiscale, c'est principalement le juge administratif qui détermine le montant des impôts fraudés. Avec le texte voté par la commission mixte paritaire, nous venons de créer, sans doute à l'insu de notre plein gré, une obligation systématique de sursis à statuer

On imagine aisément que le Conseil d'État, juge administratif suprême, ne prendrait pas très bien que le juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, fixe lui-même le montant des redressements fiscaux : comme la décision du juge pénal s'impose au juge administratif, ce dernier serait alors totalement dessaisi du contentieux fiscal d'assiette dans les dossiers transmis au pénal.

et j'attends avec impatience le décret que vous avez évoqué : vous verrez que cet article 8 est absolument inapplicable et qu'il ne donne aux justiciables aucune garantie, au contraire. La parole

l'adoption de la loi pour un État au service d'une société de confiance, qui consacre notamment le droit à l'erreur, et rétablir un certain équilibre, après la mise en oeuvre de l'échange de données entre administrations fiscales et la suppression du secret bancaire. Je ne retiendrai que deux points : la création d'une police fiscale et une avancée notable s'agissant des plateformes de commerce en ligne et de l'économie collaborative avec la reconnaissance du travail du Sénat et la publicité sur internet des sanctions fiscales pour les personnes morales.

départements. Le délai moyen entre deux vérifications peut varier en fonction de l'implantation historique des brigades départementales

l'occasion, monsieur le secrétaire d'État, de revenir sur ce point lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, à propos de l'évolution prévisible de la DGFiP au regard de l'introduction du numérique et de la dématérialisation de toutes les procédures. Je souhaite que la lutte contre la fraude fiscale reste une priorité et que, s'agissant des fautes les plus graves, les droits élargis prévus à l'article 13 du projet de loi permettent de sanctionner plus efficacement les fraudeurs, même si nous eussions pu aller plus loin.

Nous examinerons la montée en puissance dans le temps et la réalité de l'efficacité de cette police qui- je n'en doute pas -saura se montrer à la hauteur des missions qui lui seront confiées par les magistrats et trouver toute sa place. Monsieur le secrétaire d'État, je réitère mes propos de première lecture

par la commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, faire de la justice une priorité : c'est l'engagement qu'avait pris le Président de la République en 2017 devant les Français. Le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice

il est clair, il est partagé. La société française se transforme, l'État redéfinit ses missions, les services publics se modernisent, et celui de la justice n'échappe évidemment pas à ces mutations. Pour rendre le meilleur service possible aux citoyens, la justice doit se renforcer et s'adapter. Pour se renforcer, il lui faut des moyens. Or nous devons, en la matière, rattraper un retard cruel. Le Gouvernement répond donc à cette nécessité en décidant de consacrer un budget très important à la justice. Cette augmentation budgétaire est bien entendu absolument nécessaire ; elle ne saurait pourtant à elle seule suffire à relever les défis qui sont devant nous : il nous faut aussi adapter la justice aux besoins des justiciables et gagner en efficacité. Des réformes s'imposent donc. Depuis que m'a été confiée la responsabilité du ministère de la justice, je me suis évertuée à aller à la rencontre des magistrats, des greffiers, des agents, des professionnels du droit et des justiciables, partout en France. Lors de mes nombreux déplacements et au travers des échanges que j'ai pu avoir en ces occasions, j'ai été frappée par la confiance que nos concitoyens ont en l'indépendance de la justice, mais aussi par le fait qu'ils la jugent trop complexe et trop lente. Ils ont raison. Mon ambition est simple elle peut paraître modeste, mais je la crois au contraire essentielle : je souhaite que les Français se sentent protégés, écoutés, pris en considération par leur justice. J'ai la conviction profonde que la justice sera plus crédible si elle est rendue avant tout compréhensible pour les citoyens et si elle apporte des solutions en temps utile aux problèmes quotidiens qu'ils rencontrent. C'est cette conviction qui donne au projet que je vous présente ses caractéristiques propres et un contenu ambitieux. Le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice est caractérisé par trois traits

Globale, parce que le texte qui vous est présenté conjugue des moyens- c'est une loi de programmation -et des évolutions relatives aux procédures, aux méthodes et à l'organisation- c'est une loi de réforme de la justice. Concrète, cette réforme entend l'être, car elle s'appuie de manière pragmatique sur des propositions venues du terrain, dans le respect de principes indépassables, telle la garantie des droits. l'élaboration de la réforme que je vous propose, de considérations idéologiques dont notre justice a parfois trop souffert par le passé. Ma volonté est simplement de mettre en action des principes qui auront un effet direct et rapide au quotidien. C'est ce souci qui a dicté la méthode que j'ai voulu mettre en oeuvre pour construire cette loi de programmation et de réforme. Cette réforme a été construite avec les acteurs du droit et pour le justiciable. J'ai organisé une grande consultation, les chantiers de la justice, d'octobre 2017 à janvier 2018. Cette consultation m'a permis d'entendre tous les acteurs et de faire remonter des propositions issues du terrain. Des concertations ont ensuite été menées avec toutes les parties prenantes. J'ai voulu écouter les propositions, comprendre les arguments et y répondre, sans jamais abandonner mes ambitions pour la justice. Une réforme, bien entendu, suscite toujours des réactions, surtout dans notre pays. Certains expriment des craintes face au changement ; d'autres ont des aspirations nouvelles, qu'ils font valoir. Ces craintes et ces aspirations sont loin d'être toujours convergentes, selon que l'on se place du point de vue des avocats, du point de vue des magistrats ou du point de vue des élus. Pour ma part, je n'ai qu'une seule boussole : l'intérêt des justiciables, c'est-à-dire, au fond, l'intérêt général. C'est dans cet esprit que les deux projets de loi que je vous présente ont été déposés sur le bureau du Sénat. Ce choix, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, n'est pas dû au hasard : je sais le travail accompli par votre commission des lois sur ces questions.

Il s'agit, je l'ai indiqué, d'une priorité gouvernementale. Nous avons besoin de moyens pour investir et pour recruter, afin d'assurer une justice de qualité. C'est tout l'intérêt d'une loi de programmation sur cinq ans, qui offre une visibilité indispensable.

Une deuxième étape est intervenue avec le budget pour 2019 : l'augmentation de nos moyens s'accélère, avec une hausse des crédits de 4,5 % et la création de 1 300 emplois. présent projet de loi de programmation prévoit des moyens dont l'importance doit être mesurée à la hauteur de la discipline budgétaire à laquelle le Gouvernement s'astreint par ailleurs.

soit une hausse de 24 %. Cela nous permettra d'engager le recrutement de 6 500 emplois. On peut évidemment vouloir toujours plus et proposer des chiffres encore plus élevés tout est toujours possible, mais on ne peut s'abstraire d'un contexte financier et budgétaire global, et je crois qu'il ne faut pas nier le caractère positif de la mise en jeu de tels moyens au service de la justice. De l'utilisation de ces moyens, on peut attendre une amélioration des conditions de travail des magistrats et des personnels, une résorption des vacances de postes- elle a déjà commencé -et la possibilité de constituer de véritables équipes autour des magistrats. Ce budget va aussi nous permettre de passer de l'ère de l'informatique à l'ère du numérique. Il s'agit pour moi d'un élément stratégique : c'est « le » défi qu'il nous faut relever pour que la justice soit vraiment à la hauteur de l'attente des justiciables. À cette fin, nous allons engager plus d'un demi-milliard d'euros pour mener la révolution numérique. Enfin, ces moyens se déploieront naturellement dans le secteur pénitentiaire, avec la construction de 15 000 places de prison, dont 7 000 seront livrées et 8 000 engagées d'ici à 2022. Le texte comporte d'ailleurs des dispositions permettant d'accélérer la construction des établissements pénitentiaires par l'allégement de certaines procédures. Votre commission des lois les a en partie partie écartées, ce que je regrette. J'ajoute que le projet de loi de programmation prévoit la création de vingt centres d'éducation fermés. Ils constitueront l'une des réponses envisageables, parmi une gamme de propositions, à la question des jeunes mineurs délinquants.

Le contenu ambitieux du projet de loi de programmation et de réforme pour la justice se dessine autour de six axes. Le premier a trait à la procédure civile. la procédure civile. Celle-ci concerne la justice de tous les jours, de la vie quotidienne, peu spectaculaire, mais pourtant essentielle. Mon projet est simple : il faut simplifier les procédures, faciliter la vie des gens, recentrer le juge sur son coeur de métier, tout en maintenant une justice humaine, protectrice et proche des justiciables, c'est-à-dire une justice de meilleure qualité. Tel est le sens des dispositions du projet de loi.

Faciliter la vie des gens, c'est supprimer les formalités inutiles en matière de protection des majeurs vulnérables, tout en renforçant encore leurs droits fondamentaux, notamment l'exercice de leur droit de suffrage. La dématérialisation des petits litiges du quotidien est une voie à explorer et une faculté nouvelle à offrir à nos concitoyens pour plus de simplicité. La dématérialisation des injonctions de payer permettra d'obtenir une ordonnance plus rapidement. Recentrer le juge sur son coeur de métier nécessite de développer les règlements amiables des différends, comme nous le proposons. Cela suppose aussi que nous prenions en considération les outils nouveaux que sont les plateformes juridiques, mais en les encadrant avec un haut niveau de garanties pour les utilisateurs. Assurer une justice de meilleure qualité, c'est par exemple proposer d'étendre le périmètre de la représentation obligatoire par avocat. Cela s'appliquera non pas aux litiges inférieurs à 10 000 euros, mais à certains contentieux complexes, permettant d'assurer une justice de meilleure qualité. Grâce à ces mesures et à de nombreuses autres, l'expertise de l'avocat sera plus fine et mieux dirigée dans l'intérêt du client. Le travail du juge sera facilité il sera recentré sur son office et la résolution des litiges ne passera plus nécessairement par le juge, afin de pacifier et de responsabiliser la société.

Je ne partage pas les préventions de votre commission des lois quant au recours au numérique et à la dématérialisation. Ces préventions m'ont d'ailleurs étonnée, je dois l'avouer.

C'est le cas dans le projet que je porte et il ne saurait en aller autrement. Je ne souhaite pas pour ma part renoncer à l'ambition de cette réforme. Comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, le n'est pas acceptable. Mais nous en débattrons. Le deuxième axe concerne la procédure pénale. Je ne veux pas céder ici au fantasme du « grand soir » de la procédure pénale. J'ai au contraire voulu construire des solutions pratiques nées des constats issus du terrain, grâce à un travail conduit en commun avec le ministère de l'intérieur pour la phase d'enquête. La procédure pénale s'est complexifiée ces dernières années, à l'occasion de réformes qui se sont succédé, empilées, parfois sans cohérence. Cela nuit à l'action de l'autorité judiciaire et des enquêteurs. Parallèlement, la criminalité prend des formes nouvelles qui imposent davantage de réactivité et de simplicité dans l'action. Nous devons donc nous adapter pour mieux protéger les Français.

À cette fin, il faut simplifier le travail des acteurs, mieux protéger les victimes, lutter contre la délinquance du quotidien. Simplifier le travail des acteurs, qu'ils soient enquêteurs ou magistrats, est bien une priorité. C'est la raison pour laquelle je souhaite une numérisation complète des procédures. C'est aussi pour cela que le texte prévoit toute une série d'harmonisations, concernant par exemple les seuils de déclenchement de certaines procédures. Plus de clarté dans les textes et de simplicité dans les procédures, c'est naturellement une action pénale plus simple au bénéfice final des justiciables. Mieux protéger les victimes est aussi une de mes grandes préoccupations. Le dépôt de plainte en ligne constituera un réel progrès, notamment pour les victimes de violences sexuelles ou conjugales, qui hésitent parfois à franchir le seuil des commissariats pour porter plainte. Dans le même esprit,

Lutter contre la délinquance du quotidien est également une nécessité. L'instauration des amendes forfaitaires pour l'usage de stupéfiants ou l'extension de l'interdiction de comparaître constituent des exemples à cet égard. La commission des lois a approuvé cette démarche.

dans des termes souvent bien différents de ceux employés lors des réunions de travail que j'ai pu tenir avec eux, ... Comment est-ce possible ? ... pour dénoncer les atteintes qui seraient prétendument portées à la garantie des droits. J'ai d'ailleurs entendu en même temps et d'un autre côté que ce texte offrait trop de garanties, au risque d'entraver le travail des enquêteurs ... Tout cela est excessif et me semble infondé. Ce sont des postures. Je souhaite que nos débats soient l'occasion de clarifier les choses. Les garanties constitutionnelles sont bien là. J'y ai veillé. Le Conseil d'État l'a amplement confirmé dans son avis. Au renforcement des pouvoirs des enquêteurs répond le contrôle des magistrats du parquet et du siège, notamment par l'intermédiaire du juge des libertés et de la détention, sur les actes d'enquête. Je rappelle que les magistrats du parquet sont avant tout des magistrats, indépendants et garants à ce titre également de la liberté individuelle. détention, je ne crois pas que les contrôles qu'ils exercent soient de nature formelle. Par l'intervention de ce juge statutaire, la garantie des droits est bien assurée. Je dois l'avouer, je m'interroge sur la position adoptée par votre commission des lois, qui a très sensiblement modifié ce texte dans un sens qui me semble parfois éloigné des besoins réels des juridictions, des enquêteurs et des justiciables.

d'ouvrir des informations judiciaires, afin de solliciter le placement d'un suspect en détention provisoire pour éviter sa fuite, et ce alors que l'enquête est pourtant sur le point d'aboutir. Cette procédure de comparution différée pourrait épargner demain des mois de détention provisoire à ces suspects en sollicitant du juge des libertés et de la détention une détention provisoire de seulement quelques jours dans l'attente du retour des actes de procédures manquants. De même, prévoir, comme le souhaite votre commission, le droit pour les suspects d'être assistés par un avocat lors d'une perquisition créera des difficultés opérationnelles majeures pour les enquêteurs sur le terrain. Il faut être clair : sur ce plan, le texte de la commission des lois peut apparaître comme en retrait pour ce qui est de l'efficacité des enquêtes

Mais, là encore, nous en débattrons plus en détail. Le troisième axe est de redéfinir le sens et l'efficacité de la peine. Notre objectif est ici de mieux réprimer les infractions, de mieux protéger la société et de mieux réinsérer. C'est un chantier essentiel ; il doit s'envisager en lien avec le plan pénitentiaire que j'ai récemment eu l'occasion de présenter. Il faut d'abord remettre de l'ordre dans notre droit de la peine. Le postulat de base est simple : ceux qui doivent aller en prison doivent s'y rendre réellement ; ceux qui n'ont rien à y faire doivent être sanctionnés, mais d'une autre manière. C'est pourquoi je propose une nouvelle échelle des peines, considérant que toute infraction mérite sanction : en dessous d'un mois, je propose que les peines d'emprisonnement ferme soient interdites entre un et six mois, la peine s'exécutera par principe en dehors d'un établissement de détention ; entre six mois et un an, le tribunal aura la possibilité d'imposer que la peine s'exécute en détention, mais il pourra aussi orienter vers un aménagement de peine au-delà d'un an, les peines d'emprisonnement seront exécutées sans aménagement. Le seuil d'aménagement des peines d'emprisonnement sera ainsi abaissé de deux ans à un an par une modification de l'article 723-15 du code de procédure pénale. de procédure pénale. Mon objectif est de mettre fin aux emprisonnements de courte durée, très souvent inutiles, désocialisants, qui nourrissent la récidive. Mais il faut aussi assurer une exécution effective des peines prononcées. Aujourd'hui, l'inexécution des peines de prison rend incompréhensible notre justice pénale, aussi bien pour les victimes que pour les délinquants. Il faut que les peines prononcées en lieu et place de la prison soient des peines réelles, utiles et autonomes, qu'il s'agisse des travaux d'intérêt général ou de la détention à domicile sous surveillance électronique- c'est le « bracelet électronique » -, que nous proposons de

J'appelle à sortir de ces schémas tout faits, qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Je constate que votre commission des lois, si elle partage les objectifs globaux que je propose, a adopté un point de vue opérationnel différent, en particulier sur les plus courtes peines. La prison demeure pour elle un outil, une forme d'horizon pour les plus petits délits. Pour notre part, nous proposons une approche par paliers, afin de moduler davantage la réponse et de renforcer son individualisation. Elle ne souhaite pas faire du placement sous bracelet électronique une véritable peine. Ce n'est pourtant pas une commodité, mais bien une mesure coercitive, qui permet, comme l'affirmait Dominique Perben en 2004, d'« éviter la désocialisation [ ...] et le contact parfois préjudiciable avec le milieu carcéral ». Pour les courtes peines, il me semble préférable que la juridiction de jugement prononce dès le départ le placement sous bracelet électronique, le placement en semi-liberté ou un placement extérieur. Il faut assumer que ces modalités d'exécution sont plus efficaces qu'une incarcération. Si je propose par ailleurs un sursis probatoire, mêlant la contrainte pénale et le sursis avec mise à l'épreuve, c'est dans un souci d'efficacité et de souplesse, pour surmonter les difficultés rencontrées dans l'application de la peine de contrainte pénale depuis sa création. Là encore, nous partageons le même objectif, mais je crains que la peine de probation proposée par votre commission des lois ne permette pas de remédier aux lourdeurs actuelles. Nous avons là un point de divergence, que j'assume au nom de l'efficacité de la sanction et de la lutte contre la récidive. Le quatrième axe de la réforme a trait à l'évolution de l'organisation judiciaire. Il s'agit de réformer sans brutaliser. Comme je l'ai précisé devant votre commission des lois, je n'ai pas dessiné de carte ; j'ai voulu proposer une méthode. Mon projet est fondé sur deux préoccupations. D'abord, la proximité : le justiciable doit avoir un accès simple à la justice ; cela passe par une proximité physique, mais aussi par le développement du numérique. la qualité du service public de la justice : la dispersion des moyens, l'absence de spécialisation pour certains contentieux complexes ne me semblent pas être le gage d'une justice efficace. Dès l'ouverture des chantiers de la justice, j'ai affirmé qu'il n'y aurait aucune fermeture de lieux de justice. Je tiens parole. Mais il faut aussi améliorer notre organisation. Cela passe par trois évolutions principales. Le texte prévoit tout d'abord la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. L'organisation de la première instance sera ainsi plus simple pour le justiciable, qui ne connaîtra plus qu'un seul tribunal, ... Mais loin de chez Tous les sites seront maintenus, je le redis clairement, afin d'assurer une justice de proximité pour les contentieux du quotidien. J'ai également décidé, à la suite de la concertation que j'ai menée, de maintenir un juge des contentieux de la protection, qui sera chargé des tutelles, du surendettement, des crédits à la consommation et des baux d'habitation. Ce juge spécialisé statutaire traitera des contentieux ainsi identifiés comme relevant des problématiques de vulnérabilité sociale ou économique. Pour optimiser le traitement des contentieux et s'adapter au mieux à la situation de chaque ressort, les chefs de cour pourront, dans les villes où il n'existe actuellement qu'un tribunal d'instance, confier à celui-ci des contentieux autres

Une deuxième évolution concerne les départements dans lesquels il existe plusieurs tribunaux de grande instance, qui sont tous maintenus. Les chefs de cour pourront également, après concertation locale, proposer de créer dans chacun de ces tribunaux des pôles de compétences qui jugeront, pour l'ensemble du département, certains contentieux spécialisés, techniques et de faible volume. L'idée est de permettre de permettre de renforcer les compétences des magistrats là où c'est utile et d'améliorer en conséquence les délais de jugement. Enfin, le projet de loi prévoit d'expérimenter d'expérimenter dans deux régions comportant plusieurs cours d'appel l'exercice par l'une d'elles de fonctions d'animation et de coordination, ainsi que la spécialisation des contentieux selon le modèle que je viens d'évoquer. Le projet

Vous étiez partis de l'idée d'un tribunal départemental imposé par la loi. C'était une réforme qui ne me semblait pas acceptable par les territoires. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai proposé une méthode plus concrète, partant des projets territoriaux, en concertation avec les acteurs, pour conjuguer proximité et qualité de la justice.

Le cinquième axe de la réforme concerne la diversification du mode de prise en charge des mineurs délinquants. Outre la création de vingt centres éducatifs fermés, que j'ai annoncée précédemment, le texte permet de mieux préparer la sortie progressive des jeunes de ces structures, notamment le retour en famille, pour en atténuer les effets déstabilisants. Il sera aussi institué à titre expérimental une mesure éducative d'accueil de jour, troisième voie entre le placement et le milieu ouvert. Je sais le travail mené dans la Haute Assemblée par Catherine Troendlé et Michel Amiel sur ces questions, et je ne doute pas que nous évoquerons ces sujets de manière plus approfondie lors de nos débats. Le sixième axe concerne la procédure devant les juridictions administratives. Le projet de loi prévoit en effet le recrutement de juristes assistants pour renforcer les équipes autour des magistrats. Il prévoit aussi de renforcer l'exécution des décisions par des injonctions et des astreintes. Mesdames, messieurs les sénateurs, c'est bien une réforme ambitieuse que je porte. Le Gouvernement vous proposera d'ailleurs de l'enrichir, notamment par des dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, avec la création d'un parquet national spécialement dédié, dispositions qui ont été soumises à votre commission des lois. Mon objectif est à la fois simple et complexe : il s'agit de mieux servir les justiciables et la justice. Je suis certaine que nous le partageons. Sur certains Sur certains points, nous avons une approche différente. Sur d'autres, au contraire, nous nous rejoignons. Mais, ce qui nous réunit, c'est la volonté de faire que la justice de ce pays sorte enfin de l'état dans lequel elle se trouve. Cher Philippe Bas, vous vous étiez fixé comme objectif de « redresser » la justice. Je ne sais pas s'il faut la redresser, car elle me semble droite, en dépit de ses faiblesses ; ce dont je suis certaine, c'est qu'il faut la soutenir et la réformer. J'espère- je suis même convaincue -qu'ensemble nous trouverons les voies et moyens de promouvoir une réelle et belle réforme de la justice. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois,

alors même que, nous le savons tous, la surpopulation carcérale est totalement inadmissible. Exactement ! Les conditions dans lesquelles un certain nombre de détenus sont regroupés ne sont pas acceptables dans une démocratie telle que la nôtre

lois a essayé d'améliorer la rapidité et l'efficacité des procédures. Je me bornerai à citer quelques exemples à cet égard. La commission a renforcé l'encadrement des services en ligne de résolution amiable des litiges, en l'étendant aux services d'aide à la saisine des juridictions. Elle a supprimé ou restreint certaines déjudiciarisations. Elle a conservé la phase de conciliation dans les procédures de divorce contentieux. Elle a veillé à ce que la dématérialisation des procédures ne se fasse pas au détriment de l'accès au juge pour tous les justiciables. Elle a relevé le niveau de protection de la vie privée dans l'des décisions de justice, comportant l'anonymisation des magistrats. Elle a veillé

veillé à ne pas marginaliser le juge d'instruction et maintenu la collégialité des travaux de la chambre de l'instruction. La commission a garanti la présence de l'avocat lors des perquisitions. Nous avons maintenu

Marc. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et le projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions. Ce n'est pas la première fois que nous sommes saisis d'un projet de loi visant à réformer la justice. La dernière fois, c'était il y a deux ans seulement, avec la loi de modernisation de la justice du XXI siècle Alors que le diagnostic est connu depuis longtemps, de même que les pistes de réforme possibles, la situation de la justice ne s'améliore pas, car le problème de fond est bien évidemment celui des moyens. Oui, notre justice est dans un état critique aujourd'hui, car elle souffre d'un manque d'investissement prolongé, qui n'est pas du seul fait de ce gouvernement. Cette situation résulte d'une accumulation de réformes déstabilisantes souvent sous-financées, de délais de jugement qui s'allongent, d'un encombrement des juridictions civiles et pénales, d'une situation chronique de sous-effectif liée aux vacances de postes, d'un système illisible d'exécution des peines, qui conduit à ce que, souvent, la peine exécutée ne soit pas la peine prononcée,

Ce constat de la situation très dégradée de la justice, je le connais bien en ma qualité de rapporteur pour avis des crédits de l'administration pénitentiaire, tout comme la commission des lois, puisqu'il a été dressé de façon très complète dans le rapport, présenté le 4 avril 4 avril 2017, de la mission d'information sur le redressement de la justice présidée par Philippe Bas. Les différentes pistes de réforme, en dehors de la seule hausse des moyens, sont connues également. Ces dernières années, de nombreuses préconisations claires et précises sur l'organisation des juridictions, le rôle du juge ou la réforme de la procédure civile, de la procédure pénale ou du droit des peines ont été faites. Dans ces conditions, nous ne pouvons que regretter que le Gouvernement ait attendu le 20 avril 2018 pour nous présenter le projet de loi de programmation pour les années 2018 2018 à 2022 et de réforme pour la justice, ainsi que le projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions qui en est l'accessoire. Les textes qui nous sont proposés portent sur cinq grands thèmes : la programmation budgétaire, la justice civile, la procédure pénale, l'exécution des peines et l'organisation judiciaire. l'initiative de ses rapporteurs, dont je tiens à saluer à cette tribune la qualité des travaux, la commission des lois a modifié les projets de loi ordinaire et organique afin de reprendre les mesures déjà adoptées par le Sénat en octobre 2017, y compris en matière budgétaire. La commission des lois a adopté plus de 150 amendements sur ces deux textes. Ainsi, en matière budgétaire, la commission a demandé un effort plus important, à la hauteur des enjeux du redressement de la justice. En matière de justice civile, elle a amélioré l'efficacité et la rapidité des procédures, tout en veillant à la protection des personnes vulnérables, par la suppression ou l'encadrement de certaines mesures. En matière de procédure pénale, elle a été soucieuse de maintenir l'équilibre entre l'efficacité des enquêtes et la garantie des libertés, mises en danger par un renforcement excessif des prérogatives du parquet. En matière d'organisation judiciaire, la commission a clarifié la réforme, avec la création du tribunal de première instance, tout en veillant au maillage territorial et à la proximité de l'institution judiciaire. Enfin, la commission a ajouté des mesures supplémentaires de réforme, issues de ses travaux antérieurs. Je m'attarderai en particulier sur les travaux réalisés par la commission en matière d'exécution des peines, qui ont amélioré l'efficacité et la lisibilité du système, en renforçant le rôle de la juridiction de jugement et en créant une peine autonome de probation. Les règles actuelles de l'aménagement des peines conduisent à ce que les peines exécutées soient trop rarement les peines prononcées. Afin de remédier à cet état de fait, la commission a voulu donner à la juridiction de jugement la responsabilité de décider s'il y aura ou non aménagement de la peine qu'elle prononce par le juge de l'application des peines, voire de l'aménager elle-même, mais également la capacité de mieux évaluer la personnalité du condamné afin d'individualiser davantage la sanction prononcée, conformément aux conclusions de la mission d'information sur la nature Je me félicite que la commission ait ainsi restauré la crédibilité du prononcé et de l'exécution des peines, en supprimant tout examen obligatoire des peines d'emprisonnement aux fins d'aménagement. La commission a également supprimé la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en raison de la confusion qu'elle induit, et conservé le placement sous surveillance électronique. Elle a fait de la probation une peine autonome, permettant au juge de la prononcer le cas échéant en complément d'une peine d'emprisonnement. Je me réjouis enfin que la commission ait supprimé le caractère automatique de la libération sous contrainte aux deux tiers de la peine.

aucun chantier n'étant engagé à ce jour, nous pouvons malheureusement douter que même cet objectif plus modeste puisse être atteint. Madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants-République et Territoires votera en faveur de l'adoption de ces deux textes ainsi modifiés et enrichis par notre commission des lois.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues,

La nécessité d'améliorer son fonctionnement dans l'intérêt des justiciables, des citoyens et de ceux qui rendent la justice fait tout autant l'unanimité. Faire de la réforme de la justice un chantier prioritaire, c'est une volonté forte qui a été exprimée par le Président de la République et par le Premier ministre, qui en a fait d'ailleurs l'un des points essentiels de son discours de politique générale de juillet 2017. C'est la raison pour laquelle vous avez, madame la ministre, engagé dès le mois d'octobre 2017, lors des chantiers de la justice, de nombreuses consultations qui ont mené à la rédaction du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions, textes que nous examinons aujourd'hui. Des concertations ont suivi, et elles n'ont jamais cessé jusqu'à la discussion de ces deux textes au Sénat. Elles ont permis de mettre en évidence la nécessité d'améliorer la lisibilité de certaines dispositions. Je m'étonne, madame la ministre, qu'il vous soit reproché, paradoxalement, de ne pas avoir pris la mesure de l'urgence de cette réforme, d'avoir trop tardé et, dans le même temps, d'aller beaucoup trop vite en ayant engagé la procédure accélérée. Une chose est certaine : le renvoi de l'examen de ces textes du printemps 2017 à l'automne 2018 aura permis de retravailler certains points qui avaient cristallisé les mécontentements des avocats et des magistrats. Je pense, notamment, à la suppression de l'obligation de causer le divorce au moment de l'introduction de la procédure, sur laquelle la commission a pourtant décidé de revenir. Je pense également au regroupement des contentieux techniques par volume ou encore à la suppression du recours hiérarchique devant le procureur général en matière de plainte avec constitution de partie civile.

bien que perfectibles, engagent un vaste mouvement de dématérialisation, de simplification et de réorganisation du service public de la justice. Pour mettre en oeuvre cette réforme, des moyens budgétaires et humains supplémentaires ont été dégagés. projet de loi de programmation prévoyait initialement une augmentation de 24 % du budget de la justice pour les cinq prochaines années et la création de 6 500 emplois. Là encore, après que l'on eut reconnu qu'il s'agissait là d'un effort « notable », « très important », supérieur à ceux des derniers quinquennats, il a finalement été considéré qu'il n'était pas à la hauteur des enjeux du redressement de la justice.

l'argent étant le nerf de la guerre -, il existe entre nous, fort heureusement, des points de convergence, que ce soit sur les objectifs généraux ou sur des mesures concrètes, telles que la mise en place d'un mode de saisine unique en matière civile, de grande instance et l'expérimentation du tribunal criminel départemental. Néanmoins, nous vous soumettrons des amendements. Sans entrer dans le détail, je vous en présenterai brièvement les grandes lignes. Nous proposerons le rétablissement de certaines mesures, telles que la possibilité, pour le juge aux affaires familiales ou pour le parent qui y a un intérêt, de demander au procureur de la République de requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision judiciaire, une convention homologuée par le juge ou une convention de divorce par consentement mutuel enregistrée au rang des minutes d'un notaire, fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Nous demanderons également le rétablissement de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, la suppression de l'obligation de causer le divorce au moment de l'introduction de la procédure ou encore l'automaticité de la libération sous contrainte aux deux tiers de l'exécution des peines inférieures ou égales à cinq ans, sauf décision spécialement motivée du juge de l'application des peines. Compte tenu de l'importance de ces amendements, et d'autres présentés par le Gouvernement, le groupe La République en Marche conditionnera son vote à leur adoption.

Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, tribunaux engorgés, lenteur des procédures, inégalités territoriales pour les justiciables telle est la réalité de notre système judiciaire, laissé exsangue après plusieurs années pendant lesquelles maints textes sont venus restreindre l'accès au juge et les libertés individuelles. Préalablement à la rédaction de ce projet de loi, madame la ministre, vous avez mené une vaste consultation auprès des professionnels du droit, récoltant leurs doléances, leur promettant une justice « plus rapide, plus efficace et plus moderne, au service des justiciables ». La concertation a vite montré ses limites. Elle a, de fait, donné lieu à des mobilisations de professionnels de la justice Ce texte justifie, hélas ! les craintes exprimées alors par beaucoup. Encore aujourd'hui, à midi, le personnel de la justice manifestait devant le Sénat. Dématérialisation des dépôts de plainte, privatisation et déjudiciarisation de nombreuses procédures dont le juge se trouvera dépossédé au profit des notaires et de plateformes en ligne tout est bon pour réaliser des économies sur un budget de la justice déjà famélique, qui place aujourd'hui la France parmi les plus mauvais élèves de l'Union européenne en la matière. Ces dématérialisations font par ailleurs fi de nombreuses réalités humaines et sociales, notamment l'existence de déserts numériques en France. Dans la justice du « nouveau monde », la justice de proximité disparaît avec l'absorption par les tribunaux de grande instance des tribunaux d'instance, devenant des « chambres détachées Pour apaiser l'opposition des professionnels de la justice, les implantations locales seront conservées, mais elles seront vidées de leur mission ; ces tribunaux commenceront par être dévitalisés au profit d'économies substantielles et au au détriment de l'accès au droit. Sur ce dernier point, le texte prévoit le dessaisissement du juge du contentieux des pensions alimentaires, désormais traité par des organismes de droit public, les Éloigner le mineur et la famille monoparentale du juge aux affaires familiales, éloigner le majeur protégé vulnérable du juge des tutelles, voilà ce que prévoit, entre autres mesures, le volet civil de ce projet de loi C'est l'ensemble de notre justice que cette réforme met à mal : son volet pénal illustre tout autant cette réalité. Ainsi, pour ce qui concerne la lutte antiterroriste, vous faites entrer dans le droit commun un grand nombre de mesures relevant du régime d'exception.

De telles mesures sont aujourd'hui appliquées par des régimes autoritaires, ce qui devrait nous inciter à une certaine prudence. Comme le disait Montesquieu, « il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice ». Nous ne le répéterons jamais assez, l'état d'urgence est un état d'exception ; il ne saurait devenir perpétuel. Enfin, comment ne pas mentionner votre choix du « tout carcéral » en matière de politique pénitentiaire ? Beaucoup d'entre nous ont lu les rapports annuels d'Adeline Hazan, qui dénoncent un taux de surpopulation des prisons de 115 % et qui auraient dû nous inciter à conduire plutôt une politique de « déflation carcérale ça ... Comment comprendre la fin de la systématisation de l'aménagement des courtes peines, sinon comme l'expression d'une volonté de rompre avec vingt ans de politiques en faveur de la réinsertion sociale des personnes condamnées ? Prenons un autre exemple, celui de la prévention. Le Gouvernement lui préfère clairement la répression. En atteste la création d'une amende forfaitaire délictuelle à l'encontre des consommateurs de stupéfiants. Elle est dénuée de tout bon sens en matière de santé publique, alors que la consommation de cannabis est en France en nette augmentation. Madame la ministre, on reconnaît une démocratie souffrante au délitement de son système judiciaire. En instaurant une justice privée, en substituant un état d'urgence perpétuel à l'État de droit, en sacrifiant l'intérêt supérieur de l'enfant et des justiciables les plus précaires sur l'autel du libéralisme le Gouvernement semble s'engager dans une voie plutôt hasardeuse, loin des promesses de renforcement de l'efficience et de l'efficacité du système judiciaire. Notre justice mérite pourtant mieux que de se transformer en une énième branche

madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous abordons ce débat sur la réforme de la justice

Nous avions des réserves sur la question de l'exécution des peines. Le travail que nous avons accompli avec François-Noël Buffet, présenté à la commission le 12 septembre dernier, a permis d'éclaircir les choses et de donner des orientations

entend les époux, qui doivent être présents, discute avec eux des mesures provisoires et les fixe. C'est un moment important, et sa suppression procède d'une forme de déshumanisation de la justice.

pour prévenir le risque de déraillement, soit à l'éloignement géographique du milieu carcéral, par essence installé à la marge de notre société et tenu, de ce fait, à l'abri de notre regard. Tous les acteurs du droit que nous avons rencontrés pour préparer l'examen de ce projet de loi nous ont dit leur lassitude, voire leur épuisement, devant une succession de réformes n'ayant pas permis d'adapter les institutions judiciaires et pénitentiaires au besoin de justice de notre société contemporaine. Nous entendons aujourd'hui la colère des avocats et des magistrats, et nous avons toujours à l'esprit la révolte des agents pénitentiaires de l'an dernier. À l'inverse, il est rassurant de constater qu'il s'est formé un consensus au Sénat pour conduire les réformes nécessaires à la transformation de nos juridictions et au renforcement du sens de la peine. La grande qualité du rapport de MM. Détraigne et Buffet, ainsi que le travail produit en amont par MM. Buffet et Bigot, nous ont conduits à concentrer nos amendements sur quelques sujets bien ciblés que j'évoquerai plus Il est également satisfaisant d'observer que le Gouvernement a fait de ce sujet une priorité budgétaire, alors que ce projet de loi de programmation est le premier présenté pour la justice depuis 2002. Madame la garde des sceaux, nous mettons cet effort à votre crédit, et nous vous en remercions. Au-delà de l'intention positive de réforme, le champ des textes que vous soumettez aujourd'hui à notre examen est très vaste, puisqu'ils balayent le droit civil, le droit et la procédure pénale, ainsi que l'organisation judiciaire

Nous considérons que la plupart des modifications introduites par nos deux rapporteurs permettent de clarifier les logiques retenues et de lever, ici et là, quelques incohérences ou effets paradoxaux. C'est le cas notamment des modifications introduites dans le volet pénal, qui visent à restaurer le sens des peines prononcées par nos juridictions, en rapprochant les peines exécutées des peines prononcées et en réduisant l'automaticité, qui nuit à l'individualisation des décisions. Mais il ne s'agit là que du point de départ d'une réflexion qui devra être conduite sur le long terme. La marginalisation de la peine d'emprisonnement au sein de l'échelle correctionnelle des peines est également une évolution souhaitable. La commission des lois de la Haute Assemblée a également joué son rôle de protection des libertés individuelles en encadrant davantage l'extension des possibilités d'utilisation des nouvelles techniques d'enquête, le recours à la vidéo-audience et la dématérialisation des procédures.

les justiciables les plus vulnérables et à rappeler l'importance de la dimension humaine dans l'action de rendre justice. Nous ne sommes pas absolument opposés au développement de services en ligne

Nous pensons également que la crise que traverse l'institution judiciaire et le recul de la collégialité à des fins de régulation contentieuse doivent nous inciter à repenser en profondeur le rôle du juge, en relation avec les autres acteurs qui l'entourent. Le juge unique ne doit pas être un juge solitaire. Nous sommes donc très favorables au renforcement des cabinets des magistrats- sur le modèle de ce que l'on observe dans certains pays étrangers, par exemple en Italie -, qui viendrait pallier l'affaiblissement de la collégialité. On pourrait ainsi imaginer que, en plus du greffier, un magistrat soit entouré de juristes assistants, et éventuellement d'un conciliateur. La contrepartie évidente à une telle évolution doit être une meilleure valorisation des fonctions des personnels entourant le juge, greffiers comme juristes assistants. Des voies facilitant l'accès aux concours de magistrats judiciaires et administratifs doivent être prévues pour ces derniers. En outre, les propositions de nos rapporteurs visant à instaurer des formes de tutorat entre magistrats expérimentés et auditeurs de justice nous paraissent particulièrement intéressantes. la surpopulation carcérale, notre collègue Nathalie Delattre a déposé deux amendements qui, je l'espère, permettront d'engager un débat sur la place des personnes atteintes de troubles psychiques dans notre système répressif. Les représentants des familles qu'elle a rencontrés lui ont soumis des pistes pour prévenir l'incarcération de ce public aujourd'hui surreprésenté en prison. Près de 30 % des places de prison pourraient être libérées si les personnes nécessitant des soins psychiatriques étaient admises

notre plus grande crainte demeure la désertification géographique de la justice et sa concentration dans les grandes métropoles. Alors que la carte judiciaire devrait évidemment contribuer à un aménagement plus plus équilibré du territoire, elle se borne aujourd'hui à accélérer le déclin de l'activité dans nos territoires ruraux, déjà très éprouvés par le recul des services publics. Les modifications du texte introduites en commission des lois représentent à ce titre de maigres consolations, qui ne nous satisfont guère. Ces textes apportent des évolutions souhaitables, et nous les abordons de façon positive. Mais nous gardons également à l'esprit qu'ils resteront lettre morte s'ils ne s'accompagnent pas d'efforts budgétaires importants et soutenus à destination des juridictions et des services pénitentiaires, en particulier pour l'insertion et la probation. Notre groupe attend beaucoup des débats qui vont suivre.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, à la lecture de l'intitulé des deux textes qui nous sont présentés, il était légitime d'être enthousiaste : une réforme de la justice, doublée d'une programmation budgétaire pluriannuelle Le problème est effectivement principalement financier. Le tableau de bord de la justice publié par le Conseil de l'Europe classe notre pays à la vingt-troisième place en termes de pourcentage du PIB consacré à la justice.

Le Sénat prévoyait une hausse de 5 % et, surtout, la création de 13 700 emplois ... La commission a, heureusement, rétabli cette ambition.

Vous en conviendrez avec moi, la justice est un service public, une administration, certes, mais aussi et surtout l'incarnation d'un pilier de la démocratie, du « troisième pouvoir » décrit par Montesquieu, qui, malmené, mal équilibré, faute d'effectifs suffisants ou de respect vigilant de certains principes, peut broyer des vies.

La diversité, la technicité de ces deux projets de loi et le temps qui m'est imparti limitent mon propos. La discussion des articles nous permettra d'entrer dans le détail et d'approfondir. J'évoquerai tout d'abord le large mouvement de déjudiciarisation opéré par cette réforme. Nous n'avons pas d'objection de principe en la matière. Que certains actes ou certaines missions soient transférés à d'autres acteurs que l'institution judiciaire ne nous pose pas difficulté. Mais il existe malgré tout un inconvénient à cet exercice l'augmentation du coût pour le justiciable, qui perdle bénéfice de la gratuité de certains actes. Le fait que les tarifs soient réglementés limite certes le préjudice qui sera le sien, mais il ne l'annule pas : c'est là une atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi. La commission des lois a supprimé certains de ces transferts, d'autres amendements de suppression ont été déposés. Pour ce qui concerne le volet pénal, l'article 40 du projet de loi étend la compétence de la formation à juge unique du tribunal correctionnel. Depuis 1972, un nombre considérable d'affaires correctionnelles font l'objet d'un jugement rendu à juge unique, mais il s'agit des délits les plus mineurs. Le projet de loi prévoit l'introduction de près de 170 délits dans le champ de compétence du juge unique

Le tableau de bord du Conseil de l'Europe désigne nettement la surcharge des procureurs comme responsable de l'allongement des procédures. De fait, le projet de loi réduit de moitié l'augmentation des effectifs prévue par le Sénat. Sénat. En revanche, il déjudiciarise, dématérialise à tour de bras, il simplifie la procédure pénale en renforçant de manière excessive et dangereuse les prérogatives du parquet, par une réduction notable de la place du juge d'instruction. Avec ce texte, la logique inquisitoire se substitue insidieusement à la logique accusatoire La commission des lois a accompli un véritable travail de rééquilibrage. Pour n'en citer que les principaux points, elle a limité l'extension à la grande majorité des délits des techniques d'enquête intrusives dans la vie privée. Elle a veillé à ce que le juge d'instruction ne soit pas marginalisé dans la procédure pénale. Elle a maintenu la collégialité des travaux de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, garanti la présence de l'avocat lors des perquisitions, maintenu l'obligation de présentation au procureur pour la prolongation de la garde à vue, supprimé la procédure de comparution à effet différé et modéré l'extension du champ des procédures pénales transactionnelles. Accroître les pouvoirs du parquet, c'était aussi occulter le fait que, quelles que soient les compétences et la valeur professionnelle de ses membres, le parquet ne constitue pas une « autorité judiciaire » au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme fait a déjà entraîné plusieurs condamnations de la France, et la situation ne pourra s'améliorer tant que des garanties supplémentaires d'indépendance statutaire n'auront pas été apportées par une révision constitutionnelle. Le Sénat avait d'ailleurs voté cette modification dès 2013 Tant qu'une telle révision de l'article 65 de la Constitution n'aura pas été adoptée, il ne sera pas raisonnable de continuer à confier au parquet des pouvoirs toujours plus importants, surtout lorsqu'il s'agit des techniques d'enquête les plus intrusives dans la vie privée. Notre commission des lois a fait, sur ce volet du texte, un important travail, fidèle à la tradition de défense des libertés individuelles à laquelle la Haute Assemblée est si attachée. Le texte proposé par nos collègues François-Noël Buffet et Yves Détraigne permet de préserver un équilibre entre l'efficacité dans la recherche des auteurs d'infraction, d'une part, les libertés et les droits de la défense, On vient de le voir, la vague de rationalisation opérée par ce texte a préservé certains acteurs du monde judiciaire. D'autres, en revanche, ont été balayés par cette même vague : le juge d'instruction, mais aussi les jurés des cours d'assises. Cela a été rappelé, le texte prévoit la création d'un tribunal criminel qui serait compétent pour juger les personnes accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle. Je comprends l'intérêt de cette mesure par rapport à la correctionnalisation. Néanmoins, était-il nécessaire de supprimer les jurés d'assises ? Ce tribunal serait composé exclusivement de magistrats professionnels. Pourquoi vouloir se priver d'un jury citoyen ? On pourrait penser que c'est par souci d'économie, mais, si l'on s'en réfère à l'étude d'impact, il n'en est rien. On invoquera l'engorgement des cours d'assises. Mais en quoi la disparition des jurés populaires améliorerait-elle les choses ? En ces temps d'incertitude et de défiance, ne faudrait-il pas plutôt rapprocher nos concitoyens de l'institution judiciaire ? La justice n'est-elle pas rendue au nom du peuple français ? Au nom de quoi celui-ci devrait-il être écarté ? Il ne s'agit, pour le moment, que d'une expérimentation, mais on peut malgré tout s'interroger.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi de programmation pour la justice que nous examinons embrasse un grand nombre de sujets. Je me contenterai, en tant que rapporteur spécial des crédits de crédits de la mission « Justice », d'en évoquer les principaux aspects budgétaires. Je note tout d'abord avec satisfaction que le projet de loi respecte le triennal prévu par la loi de programmation des finances publiques. La trajectoire du budget du ministère de la justice est ambitieuse : elle prévoit une et 2020, contre 2,7 % pour l'ensemble des autres ministères sur la même période. Autrement dit, ce ministère prioritaire devrait bénéficier d'une augmentation très significative de ses moyens d'ici à 2020. Nous verrons dans quelques semaines dans quelle mesure le projet de loi de finances pour 2019 s'inscrit dans cette tendance. Au-delà du triennal 2018-2020,

des termes des intitulés des deux propositions de loi de notre excellent collègue Philippe Bas que le Sénat a adoptées. Il me semble toutefois qu'il convient d'être prudent : nos finances publiques s'inscrivent nécessairement dans un contexte économique et financier, et les marges de manoeuvre budgétaires dont nous disposons ne sont pas illimitées, particulièrement lorsque la croissance est dégradée. Surtout, si nous partageons tous le constat que la justice française manque cruellement de moyens, il faut également reconnaître qu'elle a besoin de se réformer. Vos projets de loi y contribuent, me direz-vous, madame la ministre. Mais je souhaiterais insister sur un domaine particulier, dans lequel il est urgent que les projets avancent réellement : je veux parler de la transformation numérique. Elle est cruciale dans une institution comme la justice. Certes, elle est en cours, mais quel chantier ! Des applications obsolètes, des réseaux indigents, des données maintes et maintes fois saisies à la main, ce qui multiplie les tâches administratives sans valeur ajoutée, ainsi que les risques d'erreur.

ne l'oubliez pas, madame la ministre ! Une part significative des moyens supplémentaires dont le ministère de la justice bénéficiera dans les prochaines années devrait prioritairement servir à doter les justiciables, comme les professionnels de la justice et du droit, d'outils numériques fiables et modernes. Vous en avez parlé, madame la garde des sceaux, comme du défi majeur devant être relevé grâce à votre réforme. Outre cet indispensable investissement dans le numérique, les moyens dégagés pourront bien sûr permettre de réduire les vacances de postes, de créer des emplois là où c'est nécessaire, et donc de diminuer les délais de jugement. Par ailleurs, ces moyens devraient permettre de rénover des établissements pénitentiaires ou d'en construire de nouveaux, pour que les conditions de détention ne soient pas indignes et que, en même temps, les conditions de travail des agents pénitentiaires soient acceptables. J'ai eu l'occasion, hier également, de rencontrer des représentants des organisations syndicales de l'administration pénitentiaire. Il semble urgent d'améliorer les conditions de travail des personnels, car créer des postes, c'est bien, mais les pourvoir, c'est mieux ! Je pense bien sûr ici aux difficultés de recrutement rencontrées par l'administration pénitentiaire, alors même que des milliers de places supplémentaires doivent être créées et qu'il faudra compenser les nombreux départs à la retraite à venir. Je pense aussi à la situation des greffes de certaines juridictions, notamment en région parisienne. De jeunes diplômés de l'École nationale des greffes renoncent au bénéfice de leur concours quand ils apprennent leur affectation au TGI de Bobigny, par exemple ! L'amélioration du fonctionnement de l'institution judiciaire passe probablement par une meilleure répartition des moyens humains sur le territoire, afin d'éviter que de jeunes professionnels, tout juste sortis d'école, ne soient affectés dans les juridictions les plus à la peine. Ce projet de loi de programmation fixe un cap.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je suis heureux de voir enfin discutés ces projets de loi qui encadrent l'action du Gouvernement en matière de justice sur la durée du quinquennat. Je suis également heureux que le Sénat ait été saisi en premier, ce qui est suffisamment rare pour être relevé. Je prends acte, par ailleurs, de la volonté du Gouvernement d'aller dans le sens d'une remise à niveau progressive- à notre sens insuffisante, il est vrai -des moyens de la justice et de réformer les procédures et les méthodes. Nous avons fait le constat de l'embolie des tribunaux et de la sous-capacité carcérale. Nous mesurons aussi les difficultés d'accès à la justice. Nous avons constaté, en outre, la stagnation aux alternatives à l'incarcération et aux peines de prison au cours des six dernières années. Nous mesurons la difficulté de la tâche, pour nous être plongés dans cette matière pendant de longs mois.

Le délai moyen d'obtention d'un jugement pour des affaires civiles est passé en deux ans de onze à douze mois. Quant aux prisons, chacun connaît la situation actuelle

du plan de construction de places de prison lancé par Michel Mercier en 2011, aucun nouveau chantier n'a été ouvert au cours des années récentes. D'où la nécessité d'un fort redressement des moyens et de réformes profondes, l'un n'allant pas sans les autres. L'idée est que la justice doit être l'objet d'une politique constante et durable, durable, au-delà des alternances, comme c'est déjà le cas depuis longtemps pour la politique de défense et la politique étrangère. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le Sénat travaille depuis plusieurs années.

à l'Assemblée nationale, préférant élaborer son propre texte, quitte à prendre davantage de temps. En effet, ce texte ne pourra pas être adopté avant 2019, alors qu'il a vocation à traiter de l'effort de redressement de la justice pour les cinq années du mandat.

2018 s'achève, et 2019 sera engagée avant l'adoption de cette loi, qui constitue donc un objet législatif singulier, à savoir une loi de programmation rétrospective

sa propre trajectoire budgétaire, adoptée par le Sénat en 2017, qui comporte une hausse des crédits de 5 % par an en moyenne, tandis que celle prévue par le Gouvernement est en deçà de 4 %.

C'est la justice des personnes les plus vulnérables qui risque ainsi d'être fragilisée. Certaines mesures transfèrent des compétences du juge à d'autres services publics : la commission les a supprimées ou strictement encadrées. D'autres vont plus loin encore en supprimant purement et simplement l'intervention du juge, sans aucun transfert de compétences judiciaire : la commission les a aussi supprimées. Dans la même veine, l'absence de toute prise en considération de la situation de l'aide juridictionnelle nous inquiète. La mission judiciaire de soutien aux plus fragiles est ainsi affaiblie.

de programmation pour le redressement de la justice que nous avions présentée visait à réformer en profondeur l'aide juridictionnelle et à assurer la pérennité de son financement. Il nous semble que l'on ne peut pas laisser de côté cette question dans une loi de programmation pour la justice. La commission veut aussi que la protection des libertés dans la procédure pénale soit renforcée par rapport à ce que prévoit le texte du Gouvernement. M. Buffet s'étant longuement exprimé sur ce point, je n'y reviens pas, mais c'est la vocation même du Sénat que d'être attentif au respect de la vie privée et à la garantie des droits fondamentaux de nos citoyens. L'efficacité des enquêtes est une cause que nous défendons dans la limite où elle ne met pas en péril les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. La commission a ainsi veillé à ne pas marginaliser le juge d'instruction et a maintenu la collégialité des travaux de la chambre d'instruction. J'en viens enfin à la politique pénitentiaire et à l'exécution des peines. La situation de nos prisons, mise en lumière par l'important mouvement social du début de cette année, n'est pas digne d'une grande démocratie. Au cours des six dernières années, le recours aux solutions alternatives à l'emprisonnement a stagné ou reculé,

ce qui aggrave les risques de récidive et l'insécurité pour la société française. La sous-capacité carcérale n'est plus traitée depuis l'abandon, en 2012, du programme de construction de places voté en 2011. Au cours de la campagne présidentielle de 2017, l'engagement de construire 15 000 places de prison en cinq ans a été pris devant les Français par plusieurs candidats, dont Emmanuel Macron. L'une des principales informations apportées par ce projet de loi, c'est

aucun site n'a été officiellement désigné pour la construction de ces 7 000 places. Par ailleurs, la réforme de l'exécution des peines nous paraît insuffisamment lisible. La commission des lois a supprimé le caractère automatique de la libération sous contrainte aux deux tiers de la peine. Madame la garde des sceaux, il y a matière à renforcer les ambitions de ce texte. Nous voulons le faire en bonne collaboration avec vous, car nous avons en réalité les mêmes objectifs. C'est ce que la commission des lois s'est attachée à faire. Je salue à cet égard le travail considérable accompli par les deux rapporteurs, qui comptent parmi les meilleurs spécialistes français de la justice. Je suis confiant dans notre capacité de progresser avec le Gouvernement dans cette voie.

que le texte que je vous soumets marginalise son rôle : au contraire, nous le recentrons sur les dossiers les plus lourds, à savoir les crimes, la criminalité organisée, les infractions économiques et financières, les atteintes graves aux personnes. Je le redis, nous entendons non pas marginaliser le juge d'instruction, mais recentrer

des motifs d'intérêt général. [ ...] Par ailleurs, il est assorti de garanties appropriées pour le demandeur que je tiens à rappeler : confidentialité de la transmission, aménagement spécial de la salle, double publicité et double procès-verbal, salle d'audience relevant du ministère de la justice et non du ministère de l'intérieur »,

vise à améliorer cette situation ; je vous remercie de l'avoir relevé. Vous avez également fait part, monsieur le sénateur, de votre intérêt pour la libération sous contrainte, qui est l'une des peines à propos desquelles la commission des lois a émis une proposition différente.

Monsieur Bigot, je vous remercie d'avoir souligné que notre plan pluriannuel est ambitieux, même si vous estimez que, sur un certain nombre d'aspects, il pourrait l'être davantage.

Vous avez absolument raison ! C'est pourquoi j'ai installé une gouvernance très serrée au sein de mon ministère sur ce sujet, avec un calendrier et des objectifs, afin que nous puissions déployer cette numérisation qui, me semble-t-il, sera l'une des conditions de l'amélioration du travail des magistrats, des personnels de greffe et également des avocats, avec lesquels nous travaillons en permanence. Vous avez soulevé

pouvoir dialoguer avec les avocats et construire avec eux un système qui soit pérenne et stable. C'est la raison pour laquelle il eût été précipité d'inscrire des dispositions définitives dans ce texte. Elles figureront sans doute dans la prochaine loi de finances, mais le financement

peuvent apparaître moins attractives que d'autres : je pense notamment à celles des surveillants pénitentiaires ou des personnels de greffe. Nous allons mettre en place, pour les surveillants pénitentiaires, des concours déconcentrés à affectation locale, ce qui permettra de résoudre cette difficulté. Nous instaurons en outre des primes de fidélisation,

La séance est reprise. Nous passons à la discussion du texte de la commission sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

cette hausse du budget, qui atteindra 1,3 milliard d'euros par an en 2022 par rapport au budget de 2018, est exprimée en euros courants, c'est-à-dire sans prendre en compte l'inflation. On sait que le Gouvernement est passé maître dans l'art de manier budget et comptabilité, mais, si l'on retient un taux d'inflation de 1,4 par an pour ces quatre années, on se rend compte que l'augmentation budgétaire réelle en 2022 s'élèvera non plus à 1,3 milliard d'euros comme annoncé, mais à seulement 900 millions d'euros. cette faible augmentation sera allouée très majoritairement aux services de l'administration pénitentiaire, et non aux services judiciaires. L'étude d'impact est explicite : cette hausse doit permettre la construction de 7 000 places de prison et l'amélioration de l'entretien du parc existant.

sur le service public de la justice rendu à nos concitoyens et sur cette justice du quotidien asphyxiée et défaillante, d'autant que le reste du texte vise dans sa globalité à éloigner davantage la justice des justiciables.

lois, d'augmenter ce budget- c'est tout à son honneur -, mais, hélas, les orientations choisies ne sont pas contestées et les carences ne sont pas comblées. En 2018, il manquait 13 000 postes pour que la France puisse rejoindre la moyenne européenne ; dès lors,

l'amélioration de l'entretien » du parc existant, « le développement des alternatives à la détention », « l'accompagnement des personnes placées sous main de justice », « le renforcement de la sécurité des établissements » pénitentiaires, « l'amélioration des conditions de travail » du personnel, l'ouverture « de vingt centres éducatifs fermés », « les moyens accordés à l'accès

corapporteur. Le présent amendement tend à rendre crédible le calendrier de la programmation budgétaire adopté par le Parlement. En effet, le Gouvernement ayant tardé à déposer et à faire examiner son projet de loi de programmation des moyens pour la justice, la loi de finances pour 2018 est déjà en cours d'exécution

Cette trajectoire intègre une réforme des peines qui a vocation à réduire le placement en détention au profit d'autres peines et donc, à terme, à diminuer le besoin en places de prison. Cette programmation permettra également, de manière plus volontariste que vous ne le proposez, de conduire un vaste plan de transformation numérique doté de 530 millions d'euros de crédits d'investissement et de 260 emplois supplémentaires. La programmation financière n'oublie pas la protection judiciaire de la jeunesse, puisqu'elle prévoit non seulement la création de vingt centres éducatifs fermés, mais également les moyens de diversifier et d'individualiser la prise en charge des mineurs par une réponse plus diversifiée et plus efficace. Enfin, ce budget donne les moyens d'une réforme globale de la justice alliant réformes des procédures civiles et de la procédure pénale, développement des modes alternatifs de règlement des litiges, adaptation de l'organisation judiciaire pour plus d'efficacité et de lisibilité, accompagnement des plus démunis par des dispositifs d'accès au droit. L'amélioration des conditions de travail dans les juridictions sera réelle. constatons d'ailleurs, après l'exécution du budget 2018 et avec le budget 2019 à venir, qu'elle commence déjà à se faire sentir grâce aux moyens prévus pour la résorption des vacances d'emploi, à la constitution des équipes entourant le magistrat que j'évoquais tout à l'heure, à un haut niveau de moyens de fonctionnement et à un effort immobilier sans précédent pour les juridictions. Pour ces raisons, le Gouvernement propose de rétablir la programmation du projet de loi initial

pour explication de vote.

Mme la ministre.

d'un amendement de coordination avec la rédaction de l'article 45 du projet de loi, qui prévoit de supprimer tout examen obligatoire des peines d'emprisonnement aux fins d'aménagement par le juge de l'application des peines et de donner à la juridiction de jugement le choix entre une exécution immédiate de la peine prononcée, un aménagement par elle-même, un mandat d'arrêt différé ou un renvoi devant le juge de l'application des peines afin de mieux préciser les modalités d'un éventuel aménagement de peine.

la conciliation comme mode de règlement apaisé et efficace des litiges. Nous sommes particulièrement engagés sur ce sujet : une campagne de recrutement de 600 conciliateurs de justice supplémentaires

à 450 euros par an et pouvant atteindre, sur autorisation des chefs de cour, 928 euros. Ce travail de recrutement de conciliateurs de justice a vocation à s'accélérer dans les prochains mois.

cet amendement tendant à supprimer la programmation du recrutement de conciliateurs de justice pour la période 2018-2022 qu'elle a introduite. L'article prévoit le recrutement de 1 500 conciliateurs de justice supplémentaires entre 2018 et 2022 par rapport à 2017, pour atteindre l'effectif de 3 420 au terme de la période. Ce besoin de recrutement a été évalué par la mission d'information du Sénat eu égard à l'extension des missions confiées aux conciliateurs de justice par la loi du 18 novembre

par coordination avec la modification de la période de programmation opérée au travers de l'amendement précédent, tend à prévoir la progression du nombre de conciliateurs de justice à compter de l'année 2019,

en fusionnant, par exemple, la médiation judiciaire et la conciliation, avec pour critère distinctif le lien avec la procédure judiciaire. L'amendement

tente de désengorger les tribunaux en encourageant le recours aux modes alternatifs de règlement des différends. Ces incitations législatives n'ont, semble-t-il, pas permis d'y parvenir.

Le présent amendement vise donc à souligner que, dès lors qu'un juge a été saisi par un justiciable et qu'il a instruit le dossier au point de considérer qu'une médiation serait possible, il pourrait permettre au justiciable en procédant lui-même à une conciliation et à l'homologation de l'accord.

opportun de faire disparaître la notion de « médiation », d'autant qu'elle est utilisée de manière générale par le droit communautaire. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

et de résolution amiable préalables aux litiges dorénavant portés devant le tribunal de grande instance, lorsque la demande n'excède pas un montant qui sera défini par décret en Conseil d'État ou lorsqu'elle a trait à un conflit de voisinage. Au choix des parties, la tentative de résolution amiable consistera en une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Votre commission des lois a supprimé cette disposition. Il me semble pourtant que les citoyens ont tout intérêt à recourir aux modes amiables de résolution des conflits. En effet, les solutions obtenues par le biais de la justice sont généralement plus pérennes, comme on peut le constater en se rendant dans un tribunal d'instance où des conciliateurs officient, ou encore dans toute autre juridiction. La variété des modes amiables qui sont admis permet de considérer que l'offre de conciliateurs de justice, de médiateurs et d'auxiliaires de justice pouvant assister les parties dans le cadre d'une convention de procédure participative sera suffisante pour que cette obligation

commission, qui a souhaité supprimer l'extension du champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des différends préalable à la saisine du juge. Si l'on ne peut que souscrire à l'objectif du Gouvernement- « développer les modes alternatifs de résolution des différends afin que afin que ne soient portées devant le juge que les affaires les plus contentieuses, pour lesquelles les parties n'ont pas pu trouver ensemble de solution amiable, et afin d'apaiser autant que possible les échanges entre les parties » -, le dispositif prévu ne nous semble pas abouti. la rédaction retenue entraînerait une restriction des modes de règlement des litiges admis, en énumérant seulement la conciliation par un conciliateur de justice, la médiation et la procédure participative, alors que les parties peuvent actuellement justifier avoir rempli leur obligation de tentative de règlement amiable de leur litige en justifiant d'autres diligences entreprises, par exemple dans le cadre d'une assurance de protection juridique, ou encore en faisant appel à un huissier de justice. En deuxième lieu, le champ d'application du dispositif nous semble imprécis. Seraient concernées par cette obligation les demandes tendant au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant que les litiges concernant les conflits de voisinage. Qu'entendre par « demandes tendant au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant » ? Que recouvre exactement la notion de « conflits de voisinage » ? Aucune définition n'en est donnée par les textes législatifs en vigueur ; la jurisprudence, quant à elle, reconnaît seulement la notion de « trouble anormal de voisinage ». En troisième lieu, le dispositif mis en place par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle est trop récent avoir produit tous ses effets et n'a pas encore été évalué. À quoi bon proposer une extension de ce dispositif, si l'on ne peut affirmer avec certitude qu'il a eu un effet positif sur le nombre de saisines des tribunaux d'instance ? En dernier lieu, le nombre de 2 400 conciliateurs nécessaire pour absorber la réforme de 2016, selon les évaluations du gouvernement de l'époque, n'a toujours pas été atteint, puisque seuls 2 021 conciliateurs sont actuellement en fonction. Or, selon le Gouvernement, s'il est difficile de quantifier les effets exacts de l'extension du dispositif, une augmentation significative de l'activité des conciliateurs est à prévoir. Il est donc prématuré, selon nous, d'envisager d'étendre le dispositif créé en 2016, sous peine de porter atteinte

dans un délai raisonnable, ne peut être jugée satisfaisante et conforte le constat que le dispositif n'est pas prêt à être étendu, faute d'un nombre suffisant de conciliateurs pour absorber le surcroît d'activité qui résulterait de cette extension. L'avis de

Je suis d'accord avec vous, et avec beaucoup de magistrats : certes, ce n'est pas dans une décision de justice qu'on trouve l'apaisement nécessaire à des conflits de voisinage ; c'est sans doute par la médiation que l'on peut espérer

c'est vieux comme le monde ! Ils ont le droit d'aller voir Saint Louis sous son chêne et de lui demander de trouver une solution. Si le magistrat n'a pas le temps, il peut désigner un médiateur,

à adopter cette mesure, qui est attendue par tout le monde. Quant au flou relevé par M. le corapporteur au sujet des litiges qui pourraient être soumis à ce type de

En effet, actuellement, afin de publier leur accord au fichier immobilier, les justiciables doivent solliciter un nouvel acte, ce qui allonge le délai de formalisation de leur accord et entraîne un coût supplémentaire pour les parties. cet amendement, de modifier l'article 710-1 du code civil afin que cette étape supplémentaire soit simplifiée pour les justiciables. En substituant la notion de « décision judiciaire » à celle de « décision juridictionnelle », une inscription directe au fichier immobilier à la suite de l'homologation du juge Cela serait particulièrement pertinent dans le cas d'un conflit de voisinage pour une petite surface de terrain, litige qui survient régulièrement en milieu rural. Or le coût de la formalité empêche souvent la résolution du conflit.

dès lors qu'ils seraient homologués par le juge. La Chancellerie a confié une mission de réflexion sur le droit de la publicité foncière au professeur Laurent Aynès. Ses propositions seront rendues publiques, si nous sommes bien informés, dans les jours qui viennent. Il n'est donc pas opportun, à nos yeux, de modifier ce droit au détour d'un amendement.

Le risque est donc de permettre la publicité d'actes entachés de vices ou difficiles à interpréter. Il apparaît donc pertinent de limiter la publicité foncière aux décisions juridictionnelles, pour lesquelles le juge opère un contrôle approfondi, et de refuser celle des décisions d'homologation, dans lesquelles il intervient de manière allégée. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

dans l'unique et seul but de désengorger les tribunaux et d'alléger la tâche des magistrats. Des sites en ligne proposeront donc désormais des services de règlement de litiges

seront bien entendu ceux qui seront les mieux servis. Voici donc le nouveau monde que l'on nous propose, dans tout ce qu'il représente de plus pernicieux pour nos services publics, qui se retrouvent dévitalisés et remplacés insidieusement par le monde de l'entreprise. Du service public défaillant au service privé efficace, il n'y a qu'un pas, que ce texte franchit. Écoutez, madame la ministre : pour notre part, ce monde, nous n'en voulons pas

qui pèseront sur l'ensemble des plateformes qui présentent leur activité sous diverses appellations : tantôt conciliation, tantôt médiation, tantôt arbitrage. Parmi les obligations que nous proposons figurent celles de diligence, de compétence, d'indépendance et d'impartialité. Nous nous donnons ainsi les moyens de garantir à nos concitoyens des services de qualité en faisant la distinction entre des opérateurs qui sont vertueux et compétents et d'autres qui ne le seraient pas. C'est tout l'objet de cet article. Le Gouvernement

Il s'agit d'un amendement de précision et de clarification rédactionnelle, concernant notamment l'usage des traitements algorithmiques de données personnelles dans le cadre des services en ligne de résolution amiable des litiges, sur la base des dispositions de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la rédaction qui résulte de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.

ni réaliser des consultations juridiques sans respecter les garanties et exigences de qualification prévues par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La certification de ces plateformes supposera une vérification du respect de ces obligations.

à cet article une référence à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, qui fixe les conditions dans lesquelles l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé peut être exercée. Cette disposition est par ailleurs rendue applicable tant aux services d'aide à la saisine en ligne qu'à ceux de résolution des litiges. La protection du périmètre du droit est une condition de la qualité des professions juridiques et judiciaires, et un gage de sécurité juridique. Nous en avons donc besoin.

sans la collaboration effective de professionnels habilités à rédiger ces actes. Afin de prémunir les futurs consommateurs de ces services contre un risque d'escroquerie et de préserver les intérêts de ces professionnels, nous proposons que les sites internet vendant de tels services de production d'actes fassent explicitement mention du nom des professionnels collaborant à leurs services, ceci dans un souci de transparence et de meilleure protection.

Mme la ministre.

des plateformes de résolution des conflits en ligne que le Gouvernement entend mettre en place. Pour assurer la confiance de nos concitoyens- je répète ce mot à dessein -, il est nécessaire d'énoncer un certain nombre d'obligations positives qui s'imposeront aux plateformes opérant dans le secteur innovant de résolution en ligne des litiges. Cependant, à la différence de la commission des lois, le Gouvernement considère que la certification doit rester

ou de santé publique, soit par le fait que la certification conditionne l'allocation de financements publics, soit par la protection des données de santé. De plus, en pratique, une certification généralisée de l'ensemble des opérateurs préalablement à la mise en service de ce dispositif paraît illusoire. À titre d'exemple, le ministère de la justice n'aura aucun moyen de contrôler un site qui serait domicilié à l'étranger et qui ne demanderait pas de certification. C'est pourquoi je vous propose, conformément au projet de loi initial, de donner un caractère facultatif à la certification des plateformes de résolution extrajudiciaire des conflits. Les utilisateurs pourront ainsi choisir, parmi les différents acteurs

des plateformes en ligne. Sur le fond, si ce caractère obligatoire peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre, il serait justifié par un objectif d'intérêt général de protection des justiciables. La résolution amiable des litiges peut s'apparenter à un démembrement d'une prérogative de puissance publique consistant à trancher des litiges, ce qui nécessite un cadre juridique précis et protecteur. Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

le recours à la conciliation ou à la médiation, y compris ce type de médiation, avant l'accès aux juges. Vous envisagez que l'obligation de se soumettre se soumettre à une médiation puisse se faire avec des organismes qui n'auraient pas besoin de demander de certification. Certes, dans l'absolu, on peut considérer qu'il appartient au justiciable de vérifier si l'organisme en ligne est certifié et quelle est sa qualité, mais vous

mauvais coton ! Je me range à l'avis du Gouvernement et de la commission sur le développement des sites de médiation. Cependant, madame le garde des sceaux, je ne comprends pas cet amendement du Gouvernement.

Il faut protéger les citoyens et ne pas donner à tous ces charlatans qui traînent aujourd'hui sur internet et qui viennent ajouter de l'escroquerie à l'escroquerie

Protégeons nos citoyens. Il y va de notre devoir, il y va du devoir de la République.

le risque du coût, c'est-à-dire le risque d'une justice inégalitaire et onéreuse pour certains, le risque de l'impartialité, du défaut de compétence et d'indépendance, que vous avez souligné, madame la ministre, la question de l'égalité de traitement et le risque de défaut de familiarité des justiciables avec ces outils numériques. L'enfer numérique est pavé de bonnes intentions. Nombre d'innovations

Il y a enfin une forme de confiance, parce que nous pensons que les arguments que nous avons fait valoir pendant le débat sur ces amendements, notamment sur le vôtre, madame la ministre, nous permettront de poursuivre le travail parlementaire et d'apporter la sécurité juridique à laquelle notre groupe est particulièrement attaché.

Il semblerait que, par extension, devant certains tribunaux paritaires, on admette que les chambres d'agriculture puissent intervenir, mais ce n'est pas automatique. Inversement, dans certains départements,

? Cet amendement tend à inclure les juristes des chambres d'agriculture dans la liste des personnes pouvant représenter une partie devant le tribunal paritaire des baux ruraux. des baux ruraux. Ce dispositif est satisfait par le droit en vigueur, qui prévoit que les parties peuvent se faire assister ou représenter dans le tribunal paritaire des baux ruraux par un membre ou salarié d'une organisation professionnelle agricole. Les chambres d'agriculture, dont nous avons d'ailleurs consulté l'assemblée permanente pour préparer notre rapport, font partie desdites organisations professionnelles agricoles aux côtés des syndicats, mais aussi des coopératives ou de tout autre groupement de personnes physiques ou morales défendant les intérêts des agriculteurs. Le code rural et de la pêche maritime, en son livre V intitulé « Organismes professionnels agricoles », définit les missions des chambres d'agriculture. Ainsi, des juristes des chambres d'agriculture interviennent fréquemment pour défendre les agriculteurs devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Dans l'objet de cet amendement, mes chers collègues,

Cette difficulté est renforcée dès lors qu'il s'agit de trouver un avocat en droit de la consommation, cette spécialisation étant rare, paraît-il. Cette proposition s'inspire d'autres matières pour lesquelles d'autres professionnels que les avocats sont déjà reconnus par la loi, notamment des représentants syndicaux ou associatifs, devant plusieurs autres juridictions spécialisées de première instance, comme les tribunaux des affaires de la sécurité sociale, les conseils de prud'hommes et les tribunaux de commerce.

ou bien en deçà d'un certain montant, cela vient d'être évoqué. À ce titre, le Gouvernement n'entend pas étendre la représentation obligatoire aux contentieux qui relevaient jusqu'à présent de la compétence du tribunal d'instance. Ainsi, les actions portant sur les crédits à la consommation, qui représentent la majorité des contentieux du droit de la consommation et qui sont, en l'état, du ressort du tribunal d'instance, ne seront pas concernées par une extension de la représentation obligatoire par avocat. Les justiciables, qui connaissent déjà une situation financière délicate, n'auront donc pas à subir un surcoût qui serait lié aux honoraires d'avocat. Pour la même raison, il ne peut être envisagé d'autoriser les associations de consommateurs à assister les parties devant le tribunal de grande instance. En effet, ces associations de consommateurs disposent déjà de la possibilité d'exercer des actions dans l'intérêt collectif des consommateurs, des actions en représentation conjointe, voire des actions de groupe. Lorsque ces actions sont engagées devant le tribunal de grande instance, ces associations sont tenues d'avoir recours au ministère d'avocat. Je n'entends pas revenir sur cet équilibre. L'objectif est d'étendre avec discernement le périmètre de la représentation par avocat, non de créer de nouvelles dérogations. J'ajoute que, en matière de droit de la consommation, le juge a l'obligation de relever d'office les moyens qui relèvent de l'ordre public, permettant ainsi d'accorder une protection aux parties, y compris lorsqu'elles ne sont ni représentées ni assistées. Par conséquent, le Gouvernement